Nadège Havet, sur l'article. Aujourd'hui, en France, lorsqu'une interruption volontaire de grossesse, ou IVG, est pratiquée, le forfait de prise en charge des frais causés est remboursé en totalité par l'assurance maladie, mais la dispense d'avance de frais, elle, n'est pas garantie dans tous les cas et pour toutes les assurées. L'absence de pratique systématique du tiers payant intégral ne permet pas, aujourd'hui, de garantir le respect du secret pour les assurées qui ont la volonté de garder leur parcours confidentiel. Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, tend à mettre fin à cette situation. Nos collègues députés ont en effet voté en faveur du tiers payant intégral systématique en cas d'interruption volontaire de grossesse, avec le souci de permettre cette confidentialité dans tous les cas de figure. Je partage cette volonté ! L'amendement adopté tendait à préciser que la prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse était protégée par le secret, afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée. Oui, les femmes doivent pouvoir y avoir recours si elles le souhaitent, sans que l'information ne soit révélée à leurs parents ou à leur conjoint ! L'amendement

Cet article est issu de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement adoptée par l'Assemblée nationale le 8 octobre dernier. Rappelons que les interruptions volontaires de grossesse sont intégralement prises en charge par l'assurance maladie et que les assurées les plus vulnérables bénéficient déjà du tiers payant assurées mineures, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, et bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Le tiers payant est, en outre, largement pratiqué dans les établissements de santé. Le dispositif proposé aurait donc essentiellement un effet sur les frais relatifs aux IVG médicamenteuses prescrites en ville. Concernant la confidentialité entourant la prise en charge des IVG, certaines dispositions permettent déjà de la garantir dans certains cas : la confidentialité est absolue pour la prise en charge des IVG des mineures sans consentement parental. Pour les assurées majeures, la feuille de soins peut être aménagée de façon à préserver la confidentialité des patientes ; le médecin de ville peut aussi les orienter vers un établissement de santé garantissant leur anonymat. Les évolutions des dispositions encadrant l'IVG, qui doivent assurer un recours effectif au droit à l'avortement, méritent un débat approfondi. Or la commission n'a pas pu apprécier pleinement la portée des dispositifs proposés, qui ont été introduits par voie d'amendement à l'Assemblée nationale nationale et qui ne relèvent pas tous du champ d'une loi de financement de la sécurité sociale. Il est préférable d'évaluer l'opportunité de ces mesures dans le cadre d'un texte spécifique. C'est pourquoi la commission présente cet amendement de suppression.

me paraissent pas rédhibitoires, et il faut s'en tenir réellement au fond : cet article améliore l'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse,

En fait, cet engagement semble avoir du mal à prendre corps. Pourtant, il faudrait qu'il devienne une réalité dans chaque territoire, et ce, finalement, quelle que soit la distance avec la maternité. Un tel engagement devrait définir dans chaque territoire les schémas d'accès aux soins de prévention,

à réduire une inégalité sexuée spécifique au système de soins en vigueur. Certains moyens de contraception, pourtant indispensables à la santé de leurs usagères, ne sont pas

de jeunes femmes qui utilisent des éponges contraceptives, des gels ou des crèmes spermicides, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.

L'application des mesures de régulation aux centres de santé, au nom d'une meilleure répartition de l'offre de soins, sur le territoire n'est pas cohérente avec la situation que nous vivons aujourd'hui

à l'opposé de l'exercice coordonné prôné par le plan Ma santé 2022 et plébiscité par les jeunes médecins, qui ne souhaitent plus exercer isolément leur métier. Pour nous, il faut encourager les aides à la création de centres de santé, qui sont également une excellente réponse en matière d'accès aux soins, car, je vous le rappelle, ces structures pratiquent le tiers payant- le secteur 1 ce qui répond aux besoins de la population, notamment des plus fragiles. La Fédération nationale des centres de santé nous a alertés sur la dangerosité d'une telle disposition : je vous encourage, mes chers collègues, à voter la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission ? Je comprends que l'introduction de ce dispositif par le Gouvernement, qui plus est par voie d'amendement, ne soit pas satisfaisante. Toutefois, cet article me semble répondre à un souci de cohérence entre les règles applicables aux professionnels de santé dans un cadre libéral ou salarié. L'article renvoie la définition des conditions et modalités à la négociation avec les fédérations de centres de santé dans le cadre de l'accord national. Je ne vois pas d'obstacle à ce que ces discussions puissent aborder cet enjeu. Même si, en l'état, le dispositif soulève des interrogations de la part de ces acteurs, il ne s'oppose pas à des discussions sur le sujet. La commission a donc émis un avis défavorable du Gouvernement ? Je tiens à rassurer Mme la sénatrice Cohen, qui souhaite supprimer un article ouvrant la possibilité aux partenaires conventionnels de négocier sur la régulation démographique au conventionnement des centres de santé, et lui rappeler la nécessité d'en discuter au préalable avec les représentants des centres de santé. Madame votre souci de prendre en compte les spécificités de l'offre de soins de ces centres de santé, car, vous l'avez dit, celle-ci n'est pas en tout point comparable avec l'offre libérale, en particulier lorsque les centres de santé sont pluriprofessionnels. C'est la raison pour laquelle cet article renvoie la déclinaison de la limitation de l'accès au conventionnement à la négociation conventionnelle, au lieu d'imposer des régulations existantes pour les professions libérales concernées. Aujourd'hui, des mesures de régulation au conventionnement existent pour certaines professions de santé libérales. Or les partenaires conventionnels ne sont pas habilités habilités à négocier sur ce sujet pour les centres de santé, et aucune régulation en zone surdotée n'est donc appliquée pour les professions concernées exerçant en centre de santé, ce qui peut aboutir à des situations incohérentes. À l'inverse, des mesures d'aide à l'installation en zone sous-dense sont proposées à la fois dans les conventions nationales monoprofessionnelles et dans l'accord national des centres de santé. Il apparaît donc justifié de permettre une négociation sur une mesure de régulation au conventionnement des centres de santé dans les zones surdotées. Enfin, si, comme vous le mentionnez, la majorité des centres de santé s'installent dans des zones sous-denses, alors la majorité des soins de santé ne sera pas concernée par une éventuelle mesure de régulation et conservera le bénéfice des éventuelles

tout à coup, on aime la régulation ... Par cet amendement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite éviter de freiner le développement des centres de santé et le déploiement de l'ensemble de leurs missions, comme le regroupement de professionnels de santé. Nous proposons également de prendre en compte dans les mesures de régulation la dimension de l'accès socio-économique aux soins, car les centres de santé, en secteur 1 essentiellement, pratiquent le tiers payant, contrairement à certaines offres libérales sur certains territoires qu'il ne s'agit pas de réguler ; on l'a bien compris. Par ailleurs, en pleine seconde vague épidémique, alors que les structures d'exercice coordonné sont pleinement mobilisées pour l'accompagnement et la prise en charge des patients, covid-19 comme non-covid-19, alors qu'elles sont impliquées dans le déploiement des stratégies de tests et qu'elles le seront encore demain dans le cadre de la stratégie vaccinale contre la covid-19, ces mesures de régulation nous paraissent précipitées et inopportunes.

Il s'agit d'un amendement de repli, qui vise à ne pas freiner le développement de centres de santé, malgré l'adoption du conventionnement des centres. Pour ce faire, nous demandons la prise en considération des caractéristiques des centres de santé dans les mesures de régulation. fondamentaux, sont les suivantes : la dimension de l'accès socio-économique aux soins, car les centres de santé sont bien souvent les dernières structures présentes sur un territoire après la disparition des professionnels libéraux, la pratique du tiers payant et l'absence de dépassements d'honoraires. Quel est l'avis de la commission

les modifications proposées tendent à s'éloigner de la cohérence avec les dispositions applicables aux professionnels libéraux, par exemple dans le cadre des maisons de santé, qui n'ont pas de régime d'exception quand ils proposent le tiers payant ou les tarifs responsables. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

défavorable. En effet, cet amendement tend à ce que les négociations conventionnelles sur un dispositif de régulation démographique au conventionnement des centres de santé se fondent sur les dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux.

Pour autant, il est nécessaire que les spécificités des centres de santé puissent être prises en compte dans les négociations et, je le répète, il n'est pas souhaitable que ces négociations soient juridiquement subordonnées aux négociations de conventions monoprofessionnelles. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement

du PLFSS pour 2019, un amendement autorisant l'expérimentation d'exercer à titre libéral en centre de santé Cela a créé une grande confusion, car cette disposition entrait en contradiction avec l'un des principes fondant l'activité des centres de santé, à savoir le salariat, qui participe de l'efficacité et de la pertinence de ce mode d'exercice regroupé et coordonné. Avant cette expérimentation, rien n'interdisait à des praticiens libéraux d'exercer dans les centres de santé, en étant salariés de ceux-ci. Comprenons-nous bien : dans ce cas, ils exercent en cabinet en tant que libéraux et, quand ils sont au centre de santé, ils exercent en tant que salariés

la commission ? Comme vous l'avez rappelé, ma chère collègue, la disposition qu'il est proposé de supprimer avait été introduite au Sénat par un amendement voté dans un précédent PLFSS. Elle nous était apparue comme une souplesse bienvenue, apportée aux praticiens dans les différents modes d'exercice libéral ou salarié. Laissons les acteurs de terrain se saisir, ou non, de cette possibilité

La ministre avait développé une argumentation centrée sur deux points. D'une part, elle avait insisté sur la nécessité de bien identifier les publics en difficulté financière, qui ne peuvent accéder au tiers payant. D'autre part, elle avait explicité la méthode qu'elle allait privilégier : rendre le tiers payant simple simple d'accès par la mise en place d'un flux unique, qui permettrait de concilier l'objectif de justice sociale et celui consistant à rendre du temps médical aux médecins. Nous avions plutôt souscrit au constat. Le tiers payant n'est pas obligatoire, par exemple, pour les pharmaciens ; pourtant, la procédure est si simple qu'elle s'est naturellement généralisée. La ministre nous avait présenté son calendrier de travail à venir, l'identification des publics prioritaires autres que ceux qui bénéficient déjà du tiers payant- par exemple, les étudiants -et du travail à engager avec les complémentaires de santé pour lever les difficultés techniques.

Mme Chantal Deseyne. Dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale, l'article 33 vise à améliorer la réforme du reste à charge zéro, en généralisant le bénéfice du tiers payant intégral pour les prestations de soins visuels, auditifs et dentaires dits « 100 % santé Si cette mesure va dans le bon sens, force est de constater qu'elle peut être améliorée pour pousser encore plus loin la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières. En effet, une enquête conduite par Ipsos en octobre 2020 montre que 20 % à 30 % des porteurs de lunettes ne bénéficient pas d'avance de frais. Cet amendement tend donc à étendre le champ de l'article 33 à l'ensemble des frais couverts par un contrat responsable.

l'avance de frais et, ainsi, de lever tout obstacle financier à l'accès à ce panier. Il oblige les organismes de complémentaire de santé proposant des contrats responsables, à compter du 1 janvier 2022, à mettre à la disposition des professionnels de santé des solutions techniques de réalisation du tiers payant qui

La rédaction de l'article 33 n'exclut pas le tiers payant pour ces équipements. Toutefois, préciser cette obligation pourrait apporter un plus aux assurés dont la complémentaire rembourse les équipements concernés.

et qu'elle peut mettre en difficulté certains professionnels de santé, qui, lorsqu'ils l'acceptent, peinent parfois à être remboursés. Il convient donc de ne pas brûler les étapes : il faut évaluer la mise en place du tiers payant sur ce panier « 100 % santé », négocié avec les différentes parties prenantes,

Sur les produits « 100 % santé », la prise en charge est intégralement garantie pour tous les assurés couverts par un contrat responsable ou par la complémentaire de santé solidaire. Le professionnel de santé connaît donc, dans tous les cas, la part prise en charge par la complémentaire de santé, ce qui ne sera pas le cas

L'article 33 vise à rendre obligatoire, à partir du 1 janvier 2022, le bénéfice du tiers payant dans les contrats responsables des complémentaires santé pour l'ensemble des prothèses optiques, dentaires et auditives.

On en compte de deux types : les lymphoedèmes secondaires, après traitement du cancer, et les lymphoedèmes primaires, liés à une anomalie. Il s'agit d'une pathologie chronique, évolutive et invalidante. Or la prise Or la prise en charge par l'assurance maladie est partielle, quels que soient les types de lymphoedèmes, et le reste à charge important pour le patient. Il peut représenter 10 % des revenus du quintile le plus pauvre de la population et 3,5 % pour les patients ayant les revenus les plus élevés. Actuellement, la prise en charge du lymphoedème comme maladie chronique ne répond donc pas aux enjeux de médicalisation de cette maladie et d'accessibilité aux traitements, et contrevient de fait à l'amélioration de la vie des patients,

plusieurs types de lymphoedèmes et leur prise en charge implique une association de traitements : physique, pharmacologique ou chirurgical. L'approche doit donc être individualisée en fonction des besoins particuliers des patients. Pour les formes primaires, qui sont plus rares, il existe un protocole national de diagnostic et de soins, qui a été élaboré par la Haute Autorité de santé, et une étude financée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui a été publiée en avril 2019.

dans le cadre de protocoles de coopération, dans des services de sécurité et de santé au travail relevant de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. Cet amendement vise à préciser les éléments à prendre en compte d'évaluation au regard des objectifs de l'expérimentation, afin d'en tirer des conclusions pertinentes en vue d'une éventuelle généralisation.

et le suivi des indicateurs mis en place relèveraient du domaine réglementaire. Madame la rapporteure, je tiens toutefois à vous rassurer : le Gouvernement entend bien se donner les moyens de suivre les effets de cette expérimentation, tant sur la couverture des obligations à la charge de ces services que sur le suivi des salariés les plus à risques et les saisonniers agricoles, ou encore sur le fonctionnement des services concernés. Ces indicateurs figurent d'ailleurs dans l'étude d'impact de cet article, sauf erreur, et seront mentionnés dans le décret d'application. Enfin, une analyse comparative avec les autres services de santé au travail en agriculture sera également

section par section, un régime d'indemnités journalières pendant les 90 premiers jours d'incapacité de travail- l'assurance invalidité pouvant prendre le relais au-delà. Ce régime est bien adapté aux professions libérales, dont les besoins en la matière sont très variables. Toutefois, aucun dispositif d'indemnités journalières n'a été mis en place par les professions libérales sur ce fondement seul le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) s'est prononcé en faveur de la mise en place de ce régime en juin 2019, mais sa démarche n'a pu aboutir. Cette absence d'un dispositif d'indemnisation des arrêts de travail a posé problème pendant la crise sanitaire. Selon l'objet de l'amendement n° 2699 déposé par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée l'État a décidé d'accorder de manière tout à fait exceptionnelle des indemnités journalières dérogatoires pour les professionnels libéraux, financées par l'assurance maladie Cette affirmation est parfaitement inexacte : seules les professions de santé ont bénéficié, à titre dérogatoire, d'indemnités journalières si elles ont été amenées à interrompre leur activité professionnelle en raison de la covid-19. Toutes les autres professions libérales ont bénéficié soit d'aménagements du règlement des cotisations sociales, soit d'aides directes financées par les sections professionnelles sur leurs fonds propres au titre de l'action sociale. Si la création d'un régime obligatoire peut se justifier, la création d'un régime unique, uniforme, n'est pas conforme à la tradition sociale des professions libérales, très attachées à leur autonomie.

Quel est l'avis de la commission ? cette logique qui tend à faire correspondre le régime créé aux réalités de chacune des professions. Je suis consciente également des craintes de voir là un nouveau régime venir alourdir les charges pour des professionnels libéraux qui ne le réclamaient pas tous et qui avaient des besoins inégaux. Rappelons que, depuis deux ans, ils avaient la possibilité de mettre ces indemnités en place, mais que toutes les caisses ne l'ont pas fait. Cependant, l'approche retenue consistant à confier ce pilotage à la CNAVPL me semble plus opportune. Renvoyer ce pilotage à chacune des sections paraît pertinent à première vue, mais risquerait, me semble-t-il, de freiner considérablement la mise en oeuvre de ce dispositif. La CNAVPL réunit bien la diversité des professions libérales et des différentes sections, que son conseil d'administration est bien chargé de proposer des adaptations. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Le problème, c'est que les régimes de sécurité sociale n'ont pas toujours une identité entre l'assiette des cotisations et le plafond retenu pour les prestations. C'est le cas, par exemple, du régime d'indemnités journalières des indépendants rattachés au régime général, qui cotisent sur deux plafonds annuels de la C'est aussi l'hypothèse retenue par le Gouvernement pour ce nouveau régime, avec une cotisation sur cinq PASS et des prestations sur trois PASS. Cette dissociation permet de répondre plus facilement, me semble-t-il, à l'impératif d'équilibre financier en assurant une redistribution. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Il convient de rappeler que, depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer des IVG par voie médicamenteuse. En revanche, les IVG instrumentales ne peuvent être réalisées que par des médecins. La pratique d'IVG instrumentales par les sages-femmes ne fait pas l'unanimité. Sur la forme, la mesure proposée, qui a trait aux compétences d'une profession de santé, est une disposition non financière, qui ne relève donc pas du champ de la loi de financement de la sécurité sociale. Pour ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet article.

Vous le savez, les sages-femmes s'investissent pleinement dans les questions de santé sexuelle et reproductive, dans une approche globale. À ce titre, elles peuvent, depuis 2016, réaliser des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.

renforcer l'accès des femmes à l'IVG en tous points du territoire et leur garantir de pouvoir choisir plus librement entre l'IVG médicamenteuse et l'IVG instrumentale, objectif que nous partageons tous, j'en suis convaincu. Cet article définit les conditions nécessaires afin d'assurer la qualité et la sécurité des soins dans le cadre de cette expérimentation, notamment en termes de formation et d'expérience

pour répondre au dernier argument de Mme la rapporteure, j'indique qu'une modification du recours à l'IVG instrumentale est à attendre en regard. Au vu des forfaits IVG,

Pour rappel, ces professionnels de santé sont habilités à pratiquer des IVG médicamenteuses depuis 2016. Le code de la santé publique garantit aux femmes la liberté de choisir entre ces deux méthodes, mais nous savons bien que, dans les faits, les IVG instrumentales représentent une part minoritaire des IVG,

Mais, mes chers collègues, puisque l'IVG médicamenteuse ou instrumentale n'est pas un acte relevant de la pathologie gynécologique, elle est, de fait, de la compétence des sages-femmes ! Cette extension des tâches, qui correspond aux objectifs du plan Ma santé 2022, est d'ailleurs très largement soutenue par nombre de médecins, qui reconnaissent les compétences des sages-femmes. Elle permettrait par ailleurs de garantir la liberté de choix de la méthode et rendrait plus accessible le recours à l'IVG partout sur le territoire, alors que plus de 130 centres IVG ont fermé en dix ans et que l'accès à celui-ci est rendu encore plus difficile en ces temps de crise sanitaire.

qu'elle devrait être réservée à des spécialistes en actes quasi chirurgicaux ? Non ! Les médecins généralistes pratiquent des IVG instrumentales ; la technique en est simple

J'ai récemment fait la connaissance d'un jeune homme que certains d'entre vous ont déjà eu, eux aussi, l'occasion de rencontrer : Hakaroa Vallé. Âgé de 15 ans, il est diabétique de type 1 et mène un combat formidable contre les discriminations que subissent les personnes diabétiques dans notre pays, notamment dans l'emploi, principalement dans la fonction publique.

deçà de 7 %, il est impossible d'être remboursé alors même qu'un tel remboursement éviterait des complications qui coûtent beaucoup plus cher à la sécurité sociale. Je tenais vraiment à aborder cette question, car cette problématique touche des milliers d'enfants et de familles en France. Nous devons tendre vers un remboursement sans condition pour les personnes insulino-dépendantes et insulino-requérantes- 500 000 Français sont concernés.

Si la volonté d'accompagner les patients atteints de pathologies chroniques dans une logique de parcours non pas seulement de santé, mais aussi de soins est partagée, le fait est que de nombreux dispositifs répondent déjà à cette finalité. L'expérimentation proposée pourrait notamment s'inscrire dans le cadre général pour l'innovation au sein du système de santé ouverte par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui avait précisément vocation à renforcer la cohérence des actions de coordination des parcours tout en renforçant leur suivi et leur évaluation. Afin de ne pas superposer les dispositifs, il est proposé de supprimer cet article.

qui viendrait s'ajouter aux dispositifs déjà mis en oeuvre pour améliorer la prévention en santé des adolescents et des jeunes adultes.

Nous avons à coeur de permettre le développement des politiques publiques en faveur de la santé sexuelle, lesquelles vont de l'éducation à la sexualité à la santé reproductive,

et dans des conditions médicales strictes, à reporter une partie de leur congé prénatal sur leur congé postnatal. Ainsi, les mères concernées pourront, sans bouleverser les dispositions actuelles et sans coût supplémentaire, disposer de plus de temps avec leur enfant après la naissance, ce qui sera favorable au développement harmonieux du lien mère-enfant. Quel

Aux mères, les soins quotidiens ; aux pères, l'éducation au savoir et la protection financière de la famille. Toutefois, cette vision patriarcale de la société a profondément changé. Aujourd'hui, ceux que l'on appelle « les nouveaux pères » cherchent à construire une paternité fondée sur la proximité la complexité affective avec leurs enfants. De plus, la naissance n'est plus uniquement une affaire de femmes : c'est un événement qui bouleverse l'existence des deux parents, du couple et de la famille. Parce qu'il répond aux attentes des familles et de très nombreux pères, l'allongement de la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est une avancée sociale majeure. Tout d'abord, la présence des deux parents pendant les premiers mois de la vie a une incidence positive durable et déterminante sur la santé et le développement des enfants. Selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui préside la commission des 1 000 premiers jours, plus le père est présent pendant la grossesse et pendant les premiers jours qui suivent la naissance, plus la mère est sécurisée et plus le bébé trouve autour de lui ce qu'il lui faut pour se développer. Nos voisins européens l'ont d'ailleurs bien compris, à l'instar de nos

Les pères ne veulent pas être traités comme des parents de seconde zone : nous devons accompagner cette évolution sociétale. Aussi, j'espère que la Haute Assemblée aura la sagesse de repousser ces amendements, pour enfin donner aux pères la place qui leur revient dans l'accueil de l'enfant.

la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, du partage des tâches ou de l'implication des deux parents, dès les premiers jours de la vie de l'enfant.

Ce doublement à vingt-huit jours, dont sept obligatoires, est un nouveau symbole du fameux « en même temps ». En avril 2019, la France faisait tout pour limiter la portée de la directive européenne relative au congé parental.

Le rapport rendu un an plus tard préconise l'extension du congé de paternité à neuf semaines et une réforme du congé parental, qui serait beaucoup mieux rémunéré Entre les grandes promesses présidentielles et la logique comptable, il a fallu trancher et, comme souvent, c'est le portefeuille qui a gagné l'arbitrage. Le congé de paternité est étendu à quatre semaines, dont une seule est obligatoire, et la réforme du congé parental est renvoyée aux calendes grecques.

essentielle, enfin, au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Seul un congé de paternité allongé dans des proportions similaires au congé de maternité permettrait de lutter contre la discrimination à l'embauche des futures mères et contre les inégalités salariales. Tant que la parentalité n'aura pas des conséquences similaires, que l'employé soit père ou mère, ces discriminations perdureront. Nous n'avons pas pu amender ce dispositif et nous le regrettons : de l'Espagne, avec ses seize semaines de congés payés, à la Suède, avec ses dix-huit mois de congés parentaux partageables, il y avait bien des modèles à suivre. à suivre. J'espère que, au-delà de la naissance, on imaginera demain dans notre pays un congé parental utilisable tout au long de la vie de l'enfant, pour l'accompagner beaucoup mieux quand le besoin s'en fait sentir !

ou ultérieurement, de manière fractionnée. Cette mesure vient soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est voulue, revendiquée, attendue par tous les parents. Depuis la création du congé de paternité, en 2002, aucun allongement n'avait été décidé. La commission des 1 000 premiers jours, qui a rendu son rapport en septembre dernier, met en avant la nécessité de renforcer ce temps parental afin de favoriser la création de liens d'attachement durables entre le second parent et l'enfant et, ainsi, d'accompagner le développement de celui-ci.

Ne nous étonnons pas, si l'on maintient cet injuste déséquilibre, que le travail professionnel des femmes soit minoré et que le principe « à travail égal, salaire égal » demeure un slogan.

aujourd'hui, l'inquiétude est grande de savoir si nos systèmes sociaux vont tenir. Le fait marquant

En effet, des absences courtes et répétées sont source de désorganisation au sein des entreprises. Certaines entreprises pourraient être confrontées à des difficultés d'aménagement des plannings si le congé était séquencé en de multiples absences de courte durée. Il est donc préférable d'aménager le congé en un fractionnement en deux blocs de périodes distinctes, en laissant la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de prévoir des règles spécifiques, le cas échéant par convention ou par accord collectif. collectif. Cet amendement vise à faciliter et à sécuriser la mise en oeuvre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant par les employeurs et par les salariés. La parole est

tendent à limiter le fractionnement à deux périodes seulement, sauf accord de l'employeur ou accord collectif plus favorable. Cette limitation me paraît restreindre la liberté du salarié de prendre les jours facultatifs de congé selon ses besoins de famille. Je ne suis pas certaine que des absences courtes soient plus déstabilisatrices pour l'entreprise que des absences longues. L'inverse peut aussi être vrai, cela dépend de la situation et des activités de l'entreprise. Je vous rappelle, en outre, que les possibilités de fractionnement

d'aligner les droits sociaux des travailleurs indépendants, qui sont souvent des travailleurs précaires, sur les droits des salariés. Ce sera l'un de nos grands chantiers à l'avenir. Il va même falloir avancer vite, car beaucoup de travailleurs indépendants sont d'abord des travailleurs précaires. Enfin, pour conclure, mais nous aurons tout le temps

Avec cet amendement, nous proposons une amélioration supplémentaire : il vise à rendre une partie du congé fractionnable au-delà d'une première période de quatorze jours calendaires. Ce fractionnement serait cautionné à un accord d'entreprise. Le fractionnement du congé de paternité et d'accueil de l'enfant permettrait ainsi d'offrir une plus grande souplesse d'organisation aux parents, tout en leur laissant la possibilité de s'impliquer plus activement à différents moments dans les semaines suivant la naissance. d'État, vous avez répondu à nos collègues députés que « l'idée du fractionnement est intéressante, mais fait actuellement l'objet de discussions avec les partenaires sociaux »,

Quel est l'avis de la commission ?

ils le feront au moment le plus opportun pour eux, pour leur enfant et pour la mère de leur enfant. De la même façon que l'on respecte la liberté des femmes

certains de mes collègues. des saisonniers, des artisans, des intermittents du spectacle, des militaires, par exemple, dont l'enfant naîtrait en pleine période d'activité professionnelle ?

Il prévoit, en outre, que cette interdiction d'emploi ne débute, le cas échéant, qu'à compter de l'issue de la période de congés payés ou de congé pour événements familiaux. Or le congé de naissance et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption font eux-mêmes partie des congés pour événements familiaux. Une lecture littérale de ce texte pourrait donc décaler l'interdiction d'emploi à l'issue du congé de naissance ou du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, ce qui est contraire à l'esprit du texte. L'évocation imprécise de l'ensemble des congés pour événements familiaux dans cet alinéa place les salariés bénéficiaires et leurs employeurs dans une insécurité juridique quant à l'application de l'interdiction d'emploi. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement vise à supprimer le caractère obligatoire du congé de naissance et des quatre premiers jours du congé de paternité.

L'amendement n° 602 rectifié vise à préciser les conditions d'interdiction d'emploi. L'article 35 prévoit que l'interdiction d'emploi du salarié pendant le congé peut débuter après la prise d'un congé payé ou pour événement familial si le salarié se trouve dans cette situation au moment où intervient la naissance. L'amendement vise à exclure de ces situations le congé de naissance et les trois jours de congé d'adoption. Or je précise que le congé d'adoption n'est pas concerné par le caractère obligatoire prévu dans le présent article. En outre, un salarié en congé d'adoption peut très bien être éligible à un congé de naissance au même moment- au titre d'un autre enfant, par exemple. Il ne me semble donc pas souhaitable d'exclure ces congés des situations permettant de différer l'interdiction d'emploi au titre du congé de naissance, car cela risque d'être trop restrictif.

les jeunes pères devraient avoir la liberté de choisir. Je respecte totalement cette approche, mais qu'en pense la mère ? Qu'en pense l'enfant ?

vaut la peine qu'on s'y attarde. L'article L. 1225-35 du code du travail ouvre le droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant au compagnon ou au partenaire de la mère, qui n'est pas le père biologique de l'enfant, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, ainsi qu'à la compagne ou épouse de la mère, dans le cadre d'un couple homosexuel. Le fait de réserver l'attribution du deuxième congé de paternité et d'accueil de l'enfant uniquement à la femme et à l'homme liés à la mère exclut donc directement de cet avantage l'homme qui vivrait maritalement avec le père, qui serait pacsé avec lui, ou qui

Cette modification aurait pourtant évité à la France le risque de se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi Maryse Carrère présente cet amendement de repli, qui vise à demander un rapport sur le caractère discriminatoire des dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail pour les couples d'hommes, et sur le coût pour les finances publiques la mise en conformité de cette disposition avec, d'une part, les prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et avec, d'autre part, la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

l'avis du Gouvernement ?

pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Un grand écart entre la durée obligatoire du congé maternité, à savoir huit semaines, dont six après l'accouchement, et celui du congé paternité, soit sept jours après la naissance de l'enfant,